des maires qui existent déjà dans la loi- il ne s'agit donc pas de créer un échelon supplémentaire -et regroupent les maires des communes d'un même bassin de vie.

des avis contraignants lorsqu'elles sont directement concernées par des délibérations du conseil métropolitain, afin de ne pas donner simplement l'illusion qu'elles sont entendues dans la métropole. Le conseil métropolitain lyonnais, du fait de son mode d'élection, ne permet pas d'assurer une représentation démocratique ni une représentation de tous les maires. Pis, nous le

de communes, qui seront en fait des opposants, voire parfois des opposants ultra-minoritaires dans certaines communes, qui siégeront au conseil métropolitain quand les maires et les membres de l'exécutif municipal n'y siégeront pas. Ce constat doit

celles-ci pouvant, en certaines circonstances, exercer un droit de veto sur les politiques de la métropole.

d'instaurer une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, ce qui est contraire à un principe constitutionnel.

le Parlement a transformé la métropole lyonnaise en collectivité territoriale. Il me semble compliqué ce soir de venir abîmer ce principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre. Néanmoins, j'y insiste, je ne me prononce pas sur l'opportunité de fond, madame la sénatrice.

: La parole est à M. Jean-Pierre Grand. Actuellement, afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre l'EPCI et les communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat. Dans sa rédaction initiale, l'article 23 du présent projet de loi rendait facultatif l'établissement de ce rapport. La rédaction adoptée par la commission des lois supprime ce rapport et transfère les modalités de mutualisation au pacte de gouvernance. Si elle peut être opportune, la mutualisation des services doit être transparente, afin de permettre aux communes membres de la contrôler. Au sujet de la transparence,

mutualisation, sans que les élus le sachent, et pas de n'importe quels services : les finances et les marchés publics ! Tout a été transféré à l'hôtel de ville de Montpellier, inaccessible aux 30 maires de la métropole.

Par ailleurs, l'absence d'obligation d'adopter un pacte de gouvernance risque de priver les conseillers communautaires des informations nécessaires sur les mutualisations en cours ou à venir. C'est totalement le cas chez nous, et ce n'est pas nouveau. Il est donc proposé de rétablir l'article L. 5211-39-1

la mutualisation est au coeur de la vocation de l'intercommunalité. Il existait précédemment un rapport de mutualisation. Au Sénat,

l'on resserre la chaîne de manière positive. Enfin, mon cher collègue, vous dites que le pacte de gouvernance n'est pas obligatoire. Certes, mais, en même temps, je ne crois pas que, dans une intercommunalité, la vôtre, il y ait

le cas d'une mutualisation de services, il y a forcément eu une délibération initiale, et de la commune et de la métropole. Sinon, c'est une juxtaposition des services dans un seul et même lieu. C'est ce que dit le droit actuel.

qu'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Par cet amendement, nous proposons d'étendre aux EPCI à fiscalité propre le référendum local, qui n'est actuellement pas prévu dans le cadre susmentionné.

Nous le voyons depuis un an avec le mouvement des « gilets jaunes », dont l'une des revendications est la participation à la décision publique. Faire participer davantage le citoyen est aussi un moyen de lui redonner envie et, par la même occasion,

1. Tout d'abord, nous souhaitons inscrire dans la loi la contribution des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon aux documents stratégiques de la métropole requis par la loi. À cette fin, la conférence métropolitaine serait obligatoirement sollicitée pour avis en amont des délibérations du conseil de la métropole sur plusieurs programmes ou schémas directeurs qui fixent les orientations générales dans les politiques publiques relevant des compétences de la métropole de Lyon, et qui sont prescrits par la loi ou les règlements.

Compte tenu des enjeux de long terme liés à cette thématique pour tout le territoire, il est prévu que la conférence métropolitaine émette un avis en amont de celui du conseil métropolitain. Ensuite, nous souhaitons inscrire dans la loi l'information des maires sur les choix budgétaires de la métropole de Lyon. À cet effet, les projets de délibération du budget primitif et ceux qui ont trait aux dotations financières aux communes situées sur le territoire de la métropole seraient soumis, uniquement pour information, à la conférence métropolitaine. Enfin, nous souhaitons modifier le nombre minimal de réunions annuelles de la conférence métropolitaine. métropolitaine. Celle-ci se réunirait au moins quatre fois par an, au lieu d'une fois au minimum, et le seuil de 50 % pour que les maires puissent en demander la convocation serait abaissé à 33 %, dans la limite de deux réunions par an, à l'instar de ce que prévoit

la liste des projets d'actes sur lesquels la conférence métropolitaine serait consultée. Vous mentionnez ainsi en obligation de consultation les projets de programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le schéma métropolitain des enseignements artistiques, le schéma d'organisation sociale et médico-sociale. S'il est légitime que les communes soient consultées sur les compétences que la métropole de Lyon exerce en leur lieu et place, votre amendement

pour l'ensemble des départements. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement.

le délai laissé à la conférence métropolitaine de la métropole de Lyon pour adopter le pacte de cohérence métropolitain, pour tenir compte de l'expérience antérieure de 2015 et du délai

M. Gilbert-Luc Devinaz. Cet amendement vise à renforcer la diversité de l'exécutif de la métropole de Lyon. Celui-ci est constitué du président, de vice-présidents, mais également d'une commission permanente, qui dispose de pouvoirs non négligeables. Jusqu'à maintenant, les conseillers membres de la commission permanente sont élus au scrutin uninominal majoritaire. Ce mode d'élection ne favorise pas la diversité et la représentativité de l'ensemble de l'assemblée. L'opposition y est notamment absente et le fait souvent remarquer. Ancien conseiller général, j'ai pu

les modalités de désignation que vous évoquez souffrent d'un déficit certain de respect de l'opposition métropolitaine. La commission émet un avis favorable. monsieur le ministre.

Je vais d'abord vous annoncer que, comme je ne bois pas de café, je ne lis pas dans le marc de café. Cependant, en prenant connaissance de la réécriture d'une partie du texte par la commission des lois,

à la volonté d'atteindre ce double objectif. Nous préférons donc demander la suppression de cet article 1 et en rester à ce qui existe aujourd'hui, même si, je l'avoue, ce n'est pas satisfaisant. Après tout, cela fait aussi partie du folklore des premières réunions des EPCI

du président de l'intercommunalité- pardon, vous savez tous cela, mais en repartant de ce constat, vous comprendrez pourquoi je suis opposé à la modification du dispositif actuel. En tout cas, je peux proposer à Mme Cukierman une piste de sortie. sortie. Ainsi, la démocratie fonctionne à plein pot et à plein tube dans l'environnement communautaire où le président de l'intercommunalité ne propose pas de liste bloquée.

une mauvaise chose, mais on change le fonctionnement même de l'intercommunalité, notamment dans le rapport entre la commune-centre, en tout cas les principales communes de l'intercommunalité, et les communes rurales.

Par définition, dans la gouvernance, il y a un moment de démocratie. Certes, il prend du temps, mais au moins, les choses se font dans la plus grande clarté. Nous savons tous que ces élections entre

par vos arguments et je vais vous exposer pourquoi. Je n'ai pas encore parlé de ma communauté de communes. Sans m'étendre sur le sujet, je dirai que j'ai moi aussi été maire et présidente d'une intercommunalité.

de coopération. Je ne doute pas que votre proposition permettrait de préserver l'intérêt des maires ruraux, mais expliquez-moi en quoi le scrutin uninominal ne provoque pas le même effet que celui que nous proposons- si tant est que celui que nous proposons ait un effet. Notre proposition vise non pas à raccourcir

de faire une liste ? J'entends votre préoccupation, monsieur le ministre, mais la proposition que vous nous faites ne garantit pas les promesses que vous nous faites.

Monsieur le ministre, je déplore votre argumentation. Il n'y a pas ici un ministre qui défendrait le monde rural et une commission des lois qui porterait atteinte aux intérêts la manière dont vous avez posé le problème est assez déplaisante, car, en réalité, votre grille d'analyse ne me paraît pas adaptée. Quand nous décidons du mode de scrutin pour l'élection du bureau, nous pensons à l'intérêt de l'intercommunalité elle-même pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion. Aucun des deux modes de scrutin ne garantit par lui-même la représentation des communes rurales. Si l'on devait choisir, on pourrait penser que, compte tenu de la nature de l'intercommunalité, le fait qu'il y ait une liste et que l'intérêt fondamental de l'exécutif de la communauté de communes soit précisément que les communes rurales y soient bien représentées protège les communes rurales contre des majorités qui se constitueraient grâce à la domination, dans le cas de figure que vous avez évoqué, des communes urbaines, dans l'intercommunalité telle que vous l'avez conçue. En réalité, nos intercommunalités sont diverses, mais aucune d'entre elles ne peut réellement fonctionner si l'on ne prend pas en compte le mieux possible toutes les communes de l'intercommunalité. En effet, la grande différence entre une intercommunalité et une municipalité- pardon de le dire, parce que c'est une évidence c'est que dans une commune de plus de 1 000 habitants, il y a souvent une majorité et une opposition. Parfois, il y a une liste unique, ce qui signifie l'absence d'opposition. Dans une communauté de communes, on ne peut pas fonctionner

monsieur le ministre, en caricaturant leur dispositif comme mettant en péril la représentation des communes rurales, que nous voulons au contraire défendre,

Soit l'on considère que la construction intercommunale doit être régie et encadrée de façon à trancher systématiquement, et de façon très claire, toutes les oppositions et tous les conflits qui pourraient voir le jour, notamment entre les villes les plus importantes et les communes les plus rurales,

parce qu'ils en ont besoin, ne serait-ce que pour des questions de ressources et de construction d'un projet. On en revient toujours au même point : je pense qu'il faut faire confiance à ces élus plutôt que de chercher à les opposer ou à encadrer leur réflexion. La

petit à petit, tout doucement, mais sûrement, on s'oriente vers une intercommunalité dont le président désignera ses vice-présidents comme un maire ses adjoints, comme un président de département ou de région ses vice-présidents. Je veux simplement que, au moment où vous vous prononcerez,

On y lit la chose suivante : « Réfléchissez également au troisième tour de l'élection, donc à vos objectifs intercommunaux. Les intercommunalités représentent un acteur crucial de la vie politique locale. C'est à ce niveau que se situent les leviers politiques les plus efficaces. Cela signifie tout simplement, monsieur le ministre, que même votre majorité reconnaît que l'enjeu politique est situé au niveau des intercommunalités

je pense très sincèrement qu'il ne faut pas introduire le scrutin de liste dans nos territoires. En outre, les gens considéreront qu'on veut politiser leurs élections.

indéniable, monsieur le rapporteur, qu'on ne fait pas la loi pour répondre à des problèmes particuliers, mais on ne la fait pas non plus en partant de bons fonctionnements particuliers. Si en Ardèche, au sein des intercommunalités, tout va très bien, tant mieux

effet, vous allez faire des vice-présidents qui n'auront pas d'autonomie. Vous allez préparer des groupes qui devront être inféodés au président de l'intercommunalité pour avoir une responsabilité. Voilà la réalité

Vous transformez, de fait, la nature de l'intercommunalité. Certes, je suis pour la politisation des débats communaux, je n'ai jamais eu peur de cette politisation, mais s'il y a politisation il doit y avoir arbitrage démocratique du peuple

la plupart des maires et, en tout cas, ceux que je connais le mieux, ceux de mon département, ne seraient pas contents, parce qu'ils auraient l'impression qu'on leur supprime encore une liberté essentielle, celle de postuler à un poste de responsabilité au sein de l'intercommunalité. J'estime donc qu'un tel changement serait tout à fait préjudiciable.

-, il faut se rappeler que le président ou la présidente de l'intercommunalité n'est pas élu au suffrage universel. Au moment même de l'élection du président, des discussions et des négociations se tiennent ; c'est aussi à l'occasion de ces négociations que se compose le bureau

Quand on est favorable à l'intercommunalité, il faut donc être défavorable à ces amendements de suppression

la gouvernance de nos intercommunalités pose effectivement problème dans beaucoup d'endroits, et le mode de désignation des vice-présidents est tout sauf anodin. tout sauf anodin. Entre la liste bloquée ou le vote par vice-président comme aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une solution idéale, mais je pense qu'il y en a une moins mauvaise.

pense qu'il vaut mieux nous en tenir au sens profond de l'intercommunalité et laisser à chacun la chance de se présenter. C'est ce que je ressens en écoutant nos collègues maires, notamment en ruralité.

cela a été souligné depuis le début de nos débats hier, l'intercommunalité est l'expression d'une volonté des communes de travailler ensemble.

et puisse présenter une liste couvrant toutes les spécificités du territoire, de la petite commune rurale au centre-bourg, voire à la commune urbaine. Mais il peut effectivement y avoir des difficultés ou des blocages Ma collègue Catherine Morin-Desailly, qui vient de s'exprimer, et moi-même connaissons bien notre département, la Seine-Maritime. Nous pourrions citer une ou deux intercommunalités dans lesquelles les choses ne se passent pas aussi bien que nous le souhaiterions.

part, je suis favorable au scrutin de liste, qui devrait permettre la recherche du consensus et donc de régler systématiquement les difficultés. Mais les difficultés peuvent exister. Aussi, monsieur le rapporteur, plutôt qu'un scrutin de liste bloquée, j'aurais souhaité que vous introduisiez la possibilité d'un scrutin de liste avec prime majoritaire.

je voudrais parler d'« équilibre ». L'équilibre n'est pas facile à trouver. Mon collègue François Patriat et moi-même faisons le tour de notre département. Nous avons des communautés « XXL » avec de toutes petites communes. Et le mot que nous entendons, cher François Patriat, c'est : « frustration ». Beaucoup de maires de petites communes ont le sentiment de ne pas avoir voix au chapitre.

Le second, applicable aux EPCI, qui sont- cela a été dit maintes fois ce soir -une construction au service des communes, fonctionne

puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote. La parité est une exigence démocratique : les femmes doivent être représentées dans les exécutifs.

est à M. le ministre. Monsieur le président Bas, vous le voyez, il n'y avait aucune malice dans mon intervention initiale.

s'il vous plaît,